Or il ne se passe pas une semaine sans que vous vous immisciez dans les discussions des partenaires sociaux, qui devaient pourtant être libres. Un jour, vous parlez de « déficit caché » ; un autre, vous imposez le retour à l’équilibre financier en 2030 ; le lendemain, vous écartez en conscience toute discussion sur l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, alors que la question est éminemment politique. Vous opérez non pas une simple révision des termes de la discussion, mais un sabotage du dispositif que vous avez vous même imaginé.

allez vous respecter vos engagements et laisser les partenaires sociaux construire une solution, sans miner le terrain des négociations ?

La première, qui est discutée très largement, est de savoir si les partenaires sociaux, organisations syndicales et représentants des entreprises,

à un retour à 62 ans. Après le 49.3 parlementaire, voici le 49.3 sur la démocratie sociale ! Ni les syndicats de salariés, ni les parlementaires, ni les citoyens n’ont le droit de proposer un retour à la retraite à 62 ans avec un financement alternatif. Sur fond de cacophonie gouvernementale, qui faut il écouter ? Les ministres dits sociaux libéraux, qui font mine de croire que tout est encore sur la table, ou les ministres clairement libéraux qui, eux, s’insurgent contre toute abrogation de cette contre réforme ? Le Premier ministre nous indique que « le contrat n’a pas changé », mais, à force de saboter les négociations, il n’y aura bientôt plus personne autour de la table pour signer un quelconque contrat. Madame la ministre

Monsieur le ministre, nous nous réjouissons que le conseil de politique nucléaire ait repris, lundi dernier, plusieurs constats et propositions de la commission d’enquête sénatoriale sur l’électricité.

d’investir dans de nouvelles technologies permettant d’exploiter le combustible usagé, afin de clore le cycle du nucléaire, c’est à dire de nous rendre indépendants de l’uranium naturel

depuis plusieurs semaines, les déclarations se succèdent pour contraindre le débat du conclave, qui devait pourtant être préservé des pressions extérieures de l’exécutif. Pour ne

en sorte que le débat soit forclos, vous méprisez une seconde fois la démocratie sociale et vous refusez la controverse sur les propositions des organisations syndicales : l’explosion des exonérations non compensées, les mesures pour une égalité salariale effective, les dispositions améliorant le taux d’emploi et le rendement des cotisations

qui, à partir du travail des partenaires sociaux, devait avoir le dernier mot ? Madame la ministre, le Gouvernement doit s’engager ici, devant nous : poursuite ou non du conclave, le Parlement sera t il saisi des propositions et paramètres qui auraient dû y être discutés ?

fois, ayez enfin le courage d’en débattre Monsieur le Premier ministre, le 18 février dernier, le Sénat a adopté, à une forte majorité, la proposition de loi qui prévoit l’interdiction des signes religieux et de l’exercice d’un culte lors des compétitions sportives. À cette occasion, le Gouvernement, par la voix de François Noël Buffet, a fermement soutenu ce texte,

que le temps passe et que le phénomène s’amplifie, monsieur le Premier ministre, ma question sera simple : quand allez vous inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ?

Je viens d’entendre votre engagement à ce que cette proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. À l’inverse de Mmes les ministres des sports et de l’éducation nationale, je rappelle l’urgence qu’il y a à légiférer sur le sujet. Il ne se passe pas un week end sans qu’un dirigeant de fédération sportive, un président de club, un éducateur, un arbitre, voire les services de police, soient confrontés à cette réalité : le sport est devenu un espace de conquête pour l’islam politique. Une large majorité de ces acteurs souhaitent

Lorsqu’on participe à une compétition, on n’a pas besoin de connaître l’appartenance religieuse ou politique de son partenaire ou de son adversaire… Que les femmes qui le portent sur les terrains de sport en aient conscience ou pas, le voile est l’instrument d’un projet politique échafaudé par les architectes d’un islam radical qui se réjouissent de l’aveuglement, de la naïveté, voire de la complicité de bon nombre de dirigeants et d’élus. Nous sommes face à un véritable enjeu de société. Ce n’est pas au sport ni à la société de s’adapter, mais bien à la religion d’évoluer. C’est la raison pour laquelle, monsieur le Premier ministre, il est urgent d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avec l’appui sans équivoque du Gouvernement. La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. et indépendants. Ma question s’adresse à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame la ministre, fermeture du golfe de Gascogne qui équivaut dans les faits à une interdiction de travailler, menace d’interdiction de certaines techniques de pêche dans les aires marines protégées, problématique de la délimitation des zones de pêche liée au Brexit, les contraintes imposées aux pêcheurs sont nombreuses. Ils doivent, comme nos agriculteurs, faire face aux nombreuses critiques ou pressions de la part de certaines organisations non gouvernementales. Ils ressentent un profond sentiment d’injustice et déplorent un paradoxe notre pêche, ce sont des emplois en mer et sur terre, c’est l’identité de nombreux territoires, et notamment celle du pays bigouden dans le Finistère. Au Guilvinec, où vous vous êtes rendue il y a quelques semaines, madame la ministre, vous avez déclaré devant les acteurs de la filière J’enrage que notre pays, qui possède la deuxième façade maritime mondiale, affiche un déficit de plus de 5 milliards d’euros dans sa balance commerciale sur la pêche pour y remédier. Nous partageons votre constat à 100 %. Depuis trente ans, la pêche française a profondément évolué : quotas stricts, progrès techniques, sélectivité accrue. Oui, ces efforts ont porté leurs fruits ! Il est aussi indispensable de renforcer ce secteur, gage de notre souveraineté alimentaire. Comment comprendre que les mareyeurs soient obligés d’importer du poisson en camion ou en avion, parce qu’ils n’ont pas la matière première pour travailler, faute de bateaux pour aller pêcher ? La logique environnementale n’est pas toujours évidente. Il y a dix jours, des pêcheurs bretons ont ainsi fait part de leur ras le bol, celui d’être pointés du doigt, d’être vus comme un problème et non comme une solution. Madame la ministre, en juin, nous accueillerons la conférence des Nations unies sur l’océan

les efforts considérables de nos pêcheurs pour mettre en place une pêche durable, de les défendre contre le phénomène de la pêche illégale, qui frappe non seulement certains territoires ultramarins, mais également

80 % des produits issus de la mer que nous consommons. C’est l’ambition que je porte dans le contrat stratégique de filière que nous avons signé avec nos pêcheurs, sous l’égide du Président de la République et du Premier ministre, lors du dernier salon de l’agriculture. Alors,

La parole est à M. Jean Luc Brault, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

auriez vous la motivation d’aller travailler vingt heures par semaine pour 95 euros par mois ? Moi, je ne l’aurais pas. Loéline, 19 ans, porteuse de trisomie 21, a ce courage. Mais on ne peut pas se résigner à ce que la ruralité aggrave le handicap. Au contraire.

Une administration qui empêche le père d’un jeune porteur de trisomie 21, avec des traits autistiques, de le représenter au téléphone. Des employeurs – et j’en sais quelque chose – qui jettent l’éponge, car trop d’interlocuteurs et trop de paperasse à remplir. Une articulation entre les différents dispositifs qui vous incite à rester à la maison.

Les personnes en situation de handicap ne veulent pas être assistées : elles veulent pouvoir s’émanciper de leur condition et œuvrer à la vie de notre cité, comme tout le monde. Les parents, les grands parents, se donnent corps et âme pour ces enfants.

ma question s’adresse à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier Runacher. La France vient de ratifier, le 5 février dernier, l’accord portant sur la protection des océans au delà des juridictions nationales. C’est un accord historique par ses objectifs et par sa méthode. Par ses objectifs, d’abord, puisqu’il porte sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité de l’océan global, en haute mer et dans les grands fonds, au delà des zones économiques exclusives. Par sa méthode, ensuite, car cet accord prévoit de compléter la Convention des Nations unies sur le droit de la mer dans le strict respect des instances déjà existantes chargées des ressources minières et de la pêche. La conférence des Nations unies sur l’océan, qui se tiendra à Nice en juin prochain, devrait, par sa dynamique, entraîner d’autres ratifications. Le gouvernement français s’est fortement impliqué dans l’élaboration de cet accord et le Parlement s’est prononcé unanimement pour sa ratification. La France, qui se veut puissance d’équilibre, dispose ici d’une occasion propice pour renforcer utilement sa diplomatie d’influence dans le monde. L’ONU, qui peine à gérer pacifiquement les contentieux de notre planète, tente cependant de jouer un fort rôle fédérateur dans la protection des océans face à des pays qui en convoitent les innombrables ressources.

Et encore faut il pouvoir maîtriser cette dernière… La mer est pourtant notre principal puits de carbone. Elle absorbe près de 30 % du CO2 que nous émettons et capte plus de 90 % de la chaleur liée au réchauffement climatique. Sans elle, le dérèglement climatique se serait emballé depuis bien longtemps.

L’annonce par Donald Trump d’une taxe de 200 % sur les vins, champagnes et spiritueux accentue une instabilité déjà préoccupante. Après les taxes de 25 % mises en place par les Américains entre 2019 et 2021, la filière, qui a toujours cherché à rester en dehors des conflits commerciaux, se retrouve une nouvelle fois en première ligne. Cette menace est une réponse aux intentions de la Commission européenne de taxer les bourbons en représailles aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium.

de l’étranger, face à ces défis, il est de notre responsabilité de protéger une filière emblématique de notre patrimoine et les milliers d’emplois qui en dépendent. Quelles actions urgentes comptez vous mettre en œuvre pour répondre à cette crise sans précédent ?

voulue par les États Unis. Concernant ce dernier point, je rappelle la position de la France : cette guerre commerciale, nous n’en voulons pas ; elle n’est bonne pour personne, à commencer

? En cas d’augmentation des droits de douane, nous l’avons dit, l’Europe doit savoir riposter, mais riposter intelligemment, c’est à dire sans mettre en danger les filières, notamment celles que vous avez évoquées. Nous dialoguons en permanence avec la Commission européenne,

Ma question s’adresse à M. le ministre d’État, ministre des outre mer. Monsieur le ministre, après le cyclone Chido, qui a dévasté notre île de Mayotte, un fort élan de solidarité s’est manifesté, notamment dans l’Hexagone. La Fondation de France évoque même un record de collecte de fonds. J’ai moi même pu mesurer la semaine dernière en Bretagne la mobilisation très importante des collectivités locales, de la petite commune à l’échelon régional. Les associations mahoraises se sont fortement mobilisées, tout comme les ONG ultramarines. Trois mois après le passage de Chido, la population mahoraise souffre en raison d’une pénurie de distribution des denrées de première nécessité, principalement l’eau.

Vous évoquez les difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire vers Mayotte. À cet égard, je salue encore une fois, comme vous l’avez fait, monsieur le sénateur, l’élan de générosité témoigné à l’égard de nos compatriotes mahorais après le passage du cyclone Chido. Aide humanitaire, denrées alimentaires, eau en bouteille : le port de Longoni est particulièrement sollicité. Son sous dimensionnement constitue, en effet, une contrainte structurelle importante. Des investissements seront nécessaires pour augmenter ses capacités et fluidifier le transport de marchandises. Dans l’immédiat, le préfet de Mayotte a réuni l’ensemble des acteurs de la chaîne portuaire et logistique, mais aussi de la grande distribution, pour fluidifier la sortie des containers et l’achalandage des commerces. Le port fonctionne de manière continue de six heures trente à quinze heures, samedi et dimanche compris. Les transporteurs travaillent également le dimanche. On ne peut pas parler d’un blocage du port. Près de 1 300 containers y sont actuellement stockés. En sortie de crise sociale, en 2024, il y en avait 7 000. La proposition de mobiliser le pouvoir de réquisition du préfet et de s’adjoindre le concours des armées pourrait être contre productive, car la réquisition s’inscrit dans un cadre juridique précis lié à l’urgence et à des impératifs d’ordre public, et réquisitionner reviendrait à interférer dans le flux logistique. J’ajoute que nos militaires sont déjà mobilisés sur des missions prioritaires : reconstitution du stock stratégique d’eau, désembâclement des ravines, Sur l’acheminement des dons, je rappelle l’importance, pour les donateurs, de prévoir, autant que faire se peut, les frais dans leur intégralité, notamment transitaires ou de manutention. Je rappelle que, à la suite de Chido, les biens destinés à l’aide aux victimes peuvent être exonérés de droits de douane et d’octroi de mer. Je rappelle également que la TVA ne s’applique pas à Mayotte.

Dans cette phase de reconstruction, soyez assuré de la pleine mobilisation de l’État aux côtés de nos compatriotes mahorais. La parole est à M. Jean François Rapin, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le ministre d’État Bruno Retailleau, vous êtes venu à deux reprises dans le Pas de Calais, sur la Côte d’Opale, pour mieux appréhender la situation migratoire sur les côtes de la Manche,

En deuxième lieu, je me suis toujours engagé à faire évoluer les Britanniques sur la question de l’attractivité du modèle anglais, qui reposait jusqu’à présent grandement sur le travail clandestin.

franco britannique, nous ne parviendrons pas à réguler cette immigration irrégulière. La frontière entre nos deux pays n’est pas seulement une frontière entre la France et le Royaume Uni : c’est une frontière extérieure européenne. puisque le Brexit a démonté l’ensemble des mécanismes d’immigration, il faut patiemment les reconstruire. De fait, 30 % de l’immigration irrégulière en Europe s’agrège

au moment de la demande, d’obtenir l’autorisation de travail et son visa pour venir en France. Je citerai également l’obligation de fournir la copie du contrat de travail signé par les deux parties. Compte tenu de la situation critique, un assouplissement vient d’être obtenu en urgence auprès de l’administration

commence dans quelques semaines, les agriculteurs du Sud Est et d’ailleurs estiment qu’il manquera cette année potentiellement 5 000 saisonniers. Madame la ministre, sommes nous certains que cet arrêté valorise le travail et protège nos agriculteurs

et même consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais, au nom de ce droit, on ne peut ni tout dire ni tout écrire. La République a ses garde fous, ses anges gardiens législatifs. Or, voilà quelques jours, un parti ayant pignon sur rue, pupitre à l’Assemblée nationale, micro ouvert dans tous les médias, a publié une affiche odieuse, directement inspirée de la propagande antisémite nazie, reprenant tous ses codes. Monsieur le ministre, cette affiche émanant non pas d’un loup solitaire ou d’un déséquilibré, mais d’un parti organisé, braconnant aux confins du champ républicain

j’ai vu cette affiche, comme beaucoup d’autres. Elle représentait deux animateurs – M. Cyril Hanouna et M. Pascal Praud. Cette affiche avait clairement des relents antisémites. Elle a été très vite retirée, certes

de l’islamisme, le brun du fascisme et le rouge sang de LFI – la France indigne, ignoble, immonde, inculte ; de ce parti qui se dit antifasciste, mais qui incarne aujourd’hui le fascisme en France… Qui sont les fachos ? … en nourrissant la bête immonde de sa pitance méphitique. Chers collègues de gauche, je vous ai entendus : réveillez vous, vous qui êtes républicains ! Brisez les chaînes de la soumission électorale qui vous lient à LFI. Amis républicains, faisons fi de LFI La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Le Gouvernement doit absolument préserver dans leur intégralité les positions actuelles des entreprises françaises sur les marchés américain et chinois.

L’implication directe du Président de la République dans des négociations bilatérales avec les États Unis est indispensable. La gravité du moment l’impose. Sur le fond,

de l’image pluriséculaire d’excellence de la France dans le monde.

des droits de douane procède de la seule volonté des États Unis. Nous l’avons dit depuis le début, la priorité est de démontrer que cette guerre commerciale n’aura que des effets

D’autres, en revanche, continuent de se voir proposer des contrats irréalistes, n’assurant aucune compétitivité, nécessitant des avances en tête exorbitantes et offrant des volumes insuffisants.

Une souveraineté territoriale bafouée, des millions de personnes déplacées, des civils massacrés et des ressources minières stratégiques : mes chers collègues, je ne vous parle pas de l’Ukraine, mais de la République démocratique du Congo (RDC) et, plus précisément, des combats qui sévissent dans le Kivu.

par l’intermédiaire de ses représentants politiques et diplomatiques, qu’a reçus notre groupe d’amitié interparlementaire France Afrique centrale. Après Goma, en janvier dernier, Bukavu est tombé en février. Aujourd’hui, les avancées du groupe rebelle armé M23, soutenu par les forces de pays voisins, exacerbent les tensions.

et la résolution de l’ONU adoptée sur l’initiative de la France, exigeant le retrait du M23 et la fin du soutien rwandais, demeure lettre morte. La France est certes intervenue, mais, de son côté, le Qatar a réuni hier les présidents rwandais et congolais pour une médiation, dans le prolongement des processus de paix de Luanda et de Nairobi.

Monsieur le ministre, pouvez vous nous rendre compte de vos actions et de celles que mène l’Union européenne pour favoriser une paix durable dans la région des Grands Lacs et, plus largement, renforcer notre coopération avec les États africains ?

pourrait provoquer l’embrasement de la région tout entière. Face à cette situation, la diplomatie française est mobilisée sur tous les fronts. La France agit tout d’abord aux Nations unies. Comme vous l’avez rappelé, nous avons fait adopter à l’unanimité du Conseil de sécurité

des mesures restrictives à l’encontre de neuf individus et d’une entité responsables de violations du droit international, en particulier du droit international humanitaire.

ont déposé une proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010 837 et de la loi n° 2010 838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis un avis favorable, voix pour et deux voix contre, sur la nomination de M. Jean Maïa aux fonctions de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes,

Michel Weber et Thierry Dulion, membres de l’Association nationale des médecins des services d’incendie et de secours (Anamnesis), « l’emploi d’une fiche d’exposition n’est pas généralisé dans l’ensemble des Sdis » et « reste une initiative locale et dépendante des moyens octroyés et de la sensibilité des responsables

Celles ci constitueront la preuve de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), ce qui permettra d’acter l’imputabilité d’un cancer à ladite exposition.

le rapport Pourny alertait sur l’absence de données épidémiologiques et préconisait « de mettre sur pied une véritable veille sanitaire des sapeurs pompiers s’appuyant sur une banque nationale de données (BND) fiable ». ». Plus de vingt ans plus tard, ni étude épidémiologique ni suivi médical coordonné n’ont été mis en œuvre. Ce manque de données s’explique notamment par le désengagement des pouvoirs publics, au fil des ans, du financement des recherches épidémiologiques, mais également par l’influence des entreprises productrices de substances potentiellement cancérogènes. J’en appelle donc aux pouvoirs publics, ainsi qu’à vous, madame la ministre, pour engager au plus vite des études épidémiologiques sérieuses.

En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a classé l’activité de sapeur pompier comme cancérogène pour l’homme et reconnu des « preuves suffisantes » pour le mésothéliome et le cancer de la vessie,

Nous invitons donc le Gouvernement à créer un tableau des maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d’extinction des incendies. Dans notre pays, ces tableaux sont établis par le Gouvernement après consultation des partenaires sociaux, selon des logiques

et les syndicats de salariés, qui luttent contre les phénomènes de sous reconnaissance. Ainsi, aujourd’hui, le cancer de la vessie et le mésothéliome, dont le lien avec l’activité de sapeur pompier et qui figurent dans les tableaux des maladies professionnelles, ne sont pas considérés comme directement imputables au service. La raison en est que la liste des travaux susceptibles de les provoquer n’inclut pas l’extinction des incendies. Il appartient donc aux sapeurs pompiers eux mêmes d’apporter la preuve du lien direct entre ces pathologies et l’exercice de leurs fonctions. C’est un comble Or nous savons que, dans le cadre de la lutte contre l’incendie, les sapeurs pompiers sont exposés à des produits de combustion cancérogènes présents dans les fumées, à l’instar des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de certains composés organiques volatils

toxiques. Les conséquences de la polyexposition demeurent de plus encore méconnues. Les expositions cumulées à des substances nocives sont en effet susceptibles de se potentialiser entre elles, avec des effets encore inconnus sur l’organisme.

attacher à les prévenir. Il existe certes une doctrine nationale de prévention, éditée par la DGSCGC, mais tous les Sdis ne se l’approprient pas de la même façon. Mieux prévenir, c’est d’abord améliorer la consultation d’aptitude à l’embauche. Il faudrait en particulier y expliquer les risques professionnels encourus, afin que les sapeurs pompiers s’acculturent eux mêmes à la nécessité de les prévenir. Chaque agent deviendrait ainsi un acteur de sa propre santé.

par une forte pression opérationnelle pour nos soldats du feu, il importe de rappeler que les sapeurs pompiers font face à des risques graves, protéiformes et, surtout, omniprésents. Je me réjouis donc que la représentation nationale se mobilise aujourd’hui afin de prendre sa part dans la protection de cette profession, dont la vocation a toujours été de protéger les autres.

de nos collègues ont notamment mis à jour un risque de sous déclaration d’ampleur des maladies professionnelles de ces agents, étayé par une observation simple : alors que le risque cancérogène des substances auxquelles ils sont quotidiennement exposés est de mieux en mieux documenté, le nombre de maladies déclarées

que le cancer de la vessie, mais également, avec des preuves plus limitées, les cancers du côlon et de la prostate, ou encore le mélanome. Selon les dernières études scientifiques, ces maladies trouveraient leur origine dans le contact quotidien des agents avec les produits de combustion des incendies, les matériaux de construction – dont l’amiante – ou encore avec les produits chimiques contenus dans les mousses anti incendie et les retardateurs de flamme.

En outre, aucun cancer professionnel n’a été détecté chez ces agents entre 2013 et 2025. Le constat d’une sous déclaration des maladies professionnelles, corroboré par ces données,

encourus empêchera d’alimenter de futurs travaux visant à perfectionner les équipements de protection ou à améliorer les protocoles de décontamination au sein des Sdis. d’information, nos collègues auteures de la proposition de loi ont expliqué cette sous déclaration par les difficultés rencontrées par les sapeurs pompiers à démontrer le lien entre leur pathologie et les missions exercées dans le cadre de leurs fonctions. En effet, hormis pour certaines maladies figurant dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale, lesquelles font en conséquence l’objet d’une présomption d’imputabilité au service, il revient à l’agent d’établir que sa pathologie est essentiellement et directement causée causée par son activité, afin d’obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle. Les difficultés de cette démonstration ne sont niées ni par les médecins ni par les Sdis. Tous reconnaissent d’ailleurs des lacunes dans le suivi de l’exposition des sapeurs

L’obligation de réaliser un relevé d’exposition à des substances nocives figure pourtant dans un décret du 5 novembre 2015. Celui ci prévoit que l’autorité territoriale réalise annuellement une synthèse relevant l’ensemble des activités potentiellement exposantes de l’agent et délivre, lorsque ce dernier quitte le Sdis, un document cumulant toutes les synthèses annuelles. Ces dossiers sont en théorie conservés pour une durée de cinquante ans. De l’aveu même des directeurs de Sdis, cependant, ces dispositions sont aujourd’hui très imparfaitement mises en œuvre. Si certains services départementaux sont proactifs et ont adopté des dispositifs de suivi très performants, d’autres sont, hélas ! en décrochage. Afin d’assurer un suivi homogène et rigoureux des risques encourus par les professionnels dans le cadre de leurs fonctions, le texte présenté par nos collègues prévoit donc d’inscrire dans la loi l’obligation pour le Sdis de réaliser une fiche d’exposition dès lors qu’un sapeur pompier a, dans le cadre de ses fonctions, été au contact d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La consécration législative de cette obligation doit susciter une réelle prise de conscience des employeurs et inciter ces derniers à se conformer aux normes en vigueur au plus vite. Elle constitue également une protection supplémentaire, car la disposition ne pourra pas être amoindrie par de futures mesures réglementaires et qu’elle fera l’objet d’une vigilance accrue de la part de la représentation nationale. Afin d’aider les directeurs de Sdis à se soumettre à cette obligation, la proposition de loi prévoit la publication de modèles nationaux de fiche d’exposition dont ils pourront se saisir afin de garantir une traçabilité, selon un modèle standardisé dans tous les départements. En effet, comme l’expliquent clairement les services départementaux, la diversité des environnements dans lesquels les sapeurs pompiers interviennent rend aujourd’hui particulièrement complexe un suivi exhaustif de leurs risques de contamination. Ces derniers dépendent en effet de la nature des combustions, du port ou non de certains équipements, ainsi que des missions confiées à l’agent au sein de l’équipe d’intervention. Au fait de ces difficultés, et certainement sensible au travail sérieux et documenté de nos collègues, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a publié, le 14 janvier dernier, des modèles nationaux de fiche d’exposition, afin d’assurer une uniformisation du suivi et,, de favoriser la reconnaissance de maladies professionnelles pour les sapeurs pompiers. La publication de ces modèles et l’adoption du présent texte constituent donc une étape afin que, partout sur le terrain, les agents se voient garantir une prise en charge dès la découverte d’une affection en lien avec leur activité. Avant de conclure, il me tient à cœur de rappeler que les dispositions proposées au travers de ce texte demeurent indissociables de réels progrès en matière de prévention. Qu’il s’agisse de réduire l’exposition au risque, notamment par les protocoles de sécurité et le port des équipements de protection, ou de détecter au plus tôt d’éventuelles pathologies par un suivi médical renforcé, la prévention est le premier rempart contre les maladies professionnelles des sapeurs pompiers. leviers que sont la prévention et la prise en charge sont les conditions d’un exercice sain et juste de missions ô combien essentielles pour nos concitoyens. Mes chers collègues, je vous demande donc d’adopter cette proposition de loi, qui constitue une garantie supplémentaire et indispensable pour la protection et la préservation de la santé des sapeurs pompiers, professionnels comme volontaires. La parole

Le Sénat a régulièrement prouvé sa grande attention aux services de lutte contre l’incendie, en s’appuyant sur l’expérience des élus locaux qui siègent dans les services départementaux d’incendie et de secours, les

comment pouvons nous mieux protéger ceux qui nous protègent ? Comment prévenir les cancers imputables à l’activité de sapeur pompier ? Si les pompiers sont habitués au danger, ils sont, hélas ! exposés à des risques moins visibles et moins directs que le feu les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui peuvent être à l’origine de maladies professionnelles, à commencer par des cancers. Si de nombreux récits de malades nous touchent et nous interpellent, nous

et pompiers volontaires à des agents toxiques. Vous proposez donc d’inscrire dans le code général de la fonction publique l’obligation, pour tous les services départementaux d’incendie et de secours, de renseigner une fiche d’exposition individuelle pour les personnels exposés, soit aux agents CMR, soit aux agents toxiques cités dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Concernant l’exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les sapeurs pompiers, comme tous les travailleurs, sont protégés par les dispositions du code du code du travail, au travers du dossier médical en santé au travail et du document unique d’évaluation des risques professionnels. L’objectif opérationnel est donc de mieux mobiliser et d’accompagner les Sdis.

Pour la santé des pompiers, nous devons et nous pouvons mieux faire. Tel est le sens de la circulaire et de la note publiées, le 14 janvier dernier, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des et fournit aux Sdis des fiches de suivi. Sa publication a été saluée par les organisations syndicales des agents des Sdis comme une avancée. Les fiches ont été élaborées dans le cadre de l’observatoire de la santé des agents des Sdis,

attentive à sa mise en œuvre, en particulier dans le cadre des évaluations par les corps d’inspection. Améliorer la traçabilité nous permettra de mieux connaître l’exposition

: nous devons actualiser les tableaux des maladies professionnelles pour qu’ils tiennent compte des maladies professionnelles et des cancers qui sont en lien avec la profession de sapeur pompier, de sorte

J’observe une grande convergence de vue entre les propositions que vous formulez et les initiatives prises par le Gouvernement pour mieux protéger ceux qui nous protègent : les soldats du feu. Je tiens donc à vous remercier de

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous nous apprêtons à voter aujourd’hui n’est pas une simple mesure bureaucratique supplémentaire. Elle n’est pas un banal ajustement technique de la réglementation du métier de sapeur pompier.

d’un engagement total, en vertu duquel on accepte d’affronter les flammes, les effondrements, les inondations, les explosions, les accidents de la route et tant d’autres situations de crise où chaque seconde compte, où chaque erreur peut être fatale. Nous connaissons tous des pompiers dans nos communes, dans nos départements. Nous avons tous vu ces hommes et ces femmes partir en intervention sans savoir s’ils reviendront indemnes. Mais ce que nous ignorons parfois, c’est que le danger ne disparaît pas une fois le feu éteint : il s’infiltre, il contamine, il ronge en silence. Les pompiers sont quotidiennement exposés à des substances hautement toxiques. Les fumées d’incendie, les particules fines, les émanations chimiques issues des matériaux brûlés contiennent des produits dont nous savons aujourd’hui qu’ils sont cancérogènes. L’amiante, les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou les dioxines sont autant de poisons invisibles qui pénètrent les poumons des pompiers, s’accumulent dans leur organisme et les condamnent, à plus ou moins long terme, à des maladies graves, souvent mortelles. Pourtant, jusqu’à présent, la reconnaissance de cette exposition et de ses conséquences sanitaires est restée insuffisante. Les pompiers tombés malades doivent encore trop souvent se battre pour faire reconnaître l’origine professionnelle de leur pathologie

L’article unique de ce texte prévoit d’ajouter dans le code général de la fonction publique un nouvel article contraignant les autorités territoriales à établir une fiche d’exposition pour chaque pompier intervenant dans des conditions présentant un risque avéré. Cette fiche, qui devra se conformer à un modèle défini par voie réglementaire, permettra de recenser précisément les substances auxquelles chaque pompier a été exposé, ainsi que les circonstances de cette exposition, et d’en assurer la traçabilité dans le temps. Il s’agit d’une avancée considérable pour nos sapeurs pompiers. Ce suivi ouvrira la voie à une reconnaissance plus rapide et plus systématique des maladies professionnelles liées à l’exposition aux agents toxiques. Il permettra d’anticiper les risques sanitaires, d’adapter les examens médicaux et les protocoles de soins, et surtout d’offrir aux sapeurs pompiers touchés par la maladie une prise en charge adaptée et digne. Cette proposition de loi constitue un premier pas, mais elle ne pourra pas être le dernier, mes chers collègues ; elle doit s’accompagner d’une réflexion beaucoup plus large sur les moyens de limiter l’exposition des pompiers à des substances dangereuses. Nous devons nous interroger sur l’amélioration des équipements de protection individuelle, sur la désinfection et le nettoyage des tenues, sur la modernisation des casernes et des véhicules pour éviter la contamination des espaces de vie. nous faut aussi nous pencher sur l’évolution des protocoles d’intervention pour réduire au maximum les risques liés aux fumées et aux produits toxiques. Aujourd’hui, ce qui est en jeu, c’est avant tout une question de justice : justice pour ces hommes et ces femmes qui, en répondant à leur vocation, en choisissant de sauver des vies, ont parfois signé leur propre condamnation, sans le savoir ; justice pour ceux qui souffrent, qui se battent contre la maladie dans un silence souvent trop pesant, loin des sirènes et des hommages ; justice, enfin, pour ceux qui ne sont plus là. Nous ne devons pas oublier que derrière ces chiffres, ces maladies professionnelles, ces cancers diagnostiqués trop tard, il y a des visages, des familles brisées, des camarades endeuillés. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nos sapeurs pompiers, professionnels ou volontaires, affrontent quotidiennement des dangers considérables. Leur engagement sans faille au service de nos concitoyens les expose à des risques graves, parmi lesquels figurent les maladies professionnelles, notamment les cancers. Lors d’une intervention, il arrive qu’ils inhalent des fumées toxiques, manipulent des substances chimiques dangereuses et évoluent dans des environnements hautement contaminés, ces expositions répétées pouvant emporter des conséquences directes sur leur santé. À ce jour, la proportion des sapeurs pompiers touchés par ces pathologies n’a, hélas ! pas fait l’objet d’une étude exhaustive en France. En juin 2022, le Circ a classé l’exposition professionnelle des sapeurs pompiers comme cancérogène pour l’homme. Ce classement repose sur des preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie, ainsi que sur des preuves limitées pour plusieurs autres cancers. cancers. Seuls deux types de cancer sont actuellement reconnus comme maladies professionnelles présumées imputables au service : le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. C’est bien peu, en comparaison de pays comme le Canada ou les États Unis, qui ont élargi cette reconnaissance. La France accuse un retard indéniable dans ce domaine. Notons aussi que les sapeurs pompiers rencontrent de grandes difficultés à faire reconnaître le lien entre leur pathologie et leur activité. En 2022, seulement trente et une maladies professionnelles ont été déclarées parmi les sapeurs pompiers professionnels, un nombre, hélas ! bien en deçà de la réalité du terrain. Face à cette situation, nos collègues Anne Marie Nédélec et Émilienne Poumirol ont déposé une proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

d’établir une fiche d’exposition dès qu’un sapeur pompier a été en contact, dans l’exercice de ses missions, avec des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou répertoriées par le code de la sécurité sociale. Afin d’assurer une mise en œuvre homogène et exhaustive de cette mesure sur l’ensemble du territoire, il prévoit également la publication de modèles de fiche d’exposition pouvant être utilisés par les autorités territoriales.

Améliorer la traçabilité des expositions permettra à nos sapeurs pompiers de mieux défendre leurs droits et d’accéder plus facilement à une reconnaissance et à une prise en charge adaptée.

Avant de conclure, je tiens à rendre hommage aux 253 000 sapeurs pompiers, professionnels et volontaires, en particulier du Sdis 59, qui, chaque jour, risquent leur vie pour sauver celle des autres. Leur engagement force le respect et mérite une reconnaissance à la hauteur de leur dévouement.

Il était donc normal de s’intéresser non seulement à leur sécurité, mais aussi à leur santé. Je rappelle qu’un observatoire de la santé des sapeurs pompiers a été créé en mai dernier, au moment où nous terminions notre mission

Elle vise à rendre obligatoire la mise au point d’un modèle national de fiche individuelle d’exposition à des facteurs de risque et à rendre systématique le renseignement d’une telle fiche après chaque intervention dangereuse, en y intégrant notamment la composition des fumées. Certes, des mesures existent pour la prévention des maladies professionnelles : médecine préventive, contrôle radiologique pulmonaire annuel ou bisannuel, etc. Depuis 2015, un suivi post professionnel a de plus été mis en place pour les pompiers qui ont été exposés à des substances cancérogènes. Il paraît néanmoins indispensable d’accroître la surveillance médicale pendant et après l’activité de sapeur pompier, y compris pour les volontaires.

La première problématique est organisationnelle. Les Sdis étant gérés de manière autonome, il n’existe pas de coordination nationale sur la prévention des risques, ce qui entraîne des disparités dans le suivi. Nous avons constaté que le remplissage des fiches d’exposition n’était ni généralisé ni toujours satisfaisant, et qu’il n’existait pas de modèle national telles fiches. Seules deux études portant sur le sujet ont été réalisées lors des dernières décennies. Publiées en 1995 et en 2012, elles concluent à une mortalité globale plus faible chez les sapeurs pompiers que dans la population générale. Cela peut paraître surprenant au regard de ce qui nous occupe aujourd’hui, mais s’explique par ce que l’on appelle le phénomène du travailleur sain : les pompiers sont généralement en meilleure santé physique que le reste de la population. Pour ce qui est de la mortalité due au cancer, la seconde étude ne notait qu’une surmortalité modérée, mais non significative, liée à certains types de cancers, alors que la première aboutissait au constat d’une mortalité supérieure pour les cancers urogénitaux, respiratoires et digestifs. La seconde problématique, qui est la principale que nous avons rencontrée pour mener à bien nos travaux, tient à l’absence de données épidémiologiques suffisamment précises et exploitables. Cette difficulté est accrue dans un système de protection civile comme le nôtre, où interviennent massivement les sapeurs pompiers volontaires, dans la mesure où ces derniers exercent par ailleurs une activité professionnelle susceptible de les exposer à des agents cancérogènes ou mutagènes. Un suivi fin des expositions lors des interventions se révèle donc d’autant plus nécessaire. Si le lien entre l’exposition à des fumées potentiellement toxiques et le développement de certains cancers peut paraître intuitif, notre pays ne dispose pas de données fiables à exploiter.

: les données sont souvent partielles et les missions des pompiers comme le cadre d’intervention ne sont pas totalement analogues d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre.

De même, la reconnaissance de ces maladies imputables au service diffère dans le monde, la France étant par exemple la seule à reconnaître le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. À titre de comparaison, au Canada, neuf cancers sont reconnus imputables au service au Québec et dix neuf en Ontario. L’absence de données fiables demeure donc un véritable frein.

renforçant le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles des sapeurs pompiers. Je tiens à saluer le travail engagé par les ministères de l’intérieur et du travail qui, conscients des enjeux,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chaque jour, nos 253 000 sapeurs pompiers professionnels et volontaires sont en première ligne pour protéger nos concitoyens. Face aux flammes, aux émanations toxiques, aux substances dangereuses, ils risquent leur vie, mais aussi, et peut être plus insidieusement encore, leur santé. Si leur engagement est perçu comme héroïque, n’oublions jamais qu’ils sont avant tout des femmes, des hommes, des travailleurs qui méritent la reconnaissance et la solidarité de la Nation, lesquelles doivent se traduire par des actes concrets. Tel est précisément l’objet du texte qui nous réunit aujourd’hui. Les risques auxquels les sapeurs pompiers sont confrontés sont multiples

a classé leur activité comme cancérogène pour l’homme, mettant en évidence des liens directs avec certains cancers, notamment le mésothéliome et le cancer de la En dépit de cette réalité accablante, la reconnaissance des maladies professionnelles demeure un parcours du combattant pour ceux qui en sont victimes. Ainsi, en 2023, seuls vingt quatre cas de maladies professionnelles ont été déclarés chez les sapeurs pompiers, soit un taux de 0,55 % de sinistralité

Les raisons en sont connues : difficulté à obtenir la preuve de l’exposition, manque de traçabilité des interventions et, surtout, absence de reconnaissance automatique de certaines pathologies comme étant imputables au service. Aujourd’hui encore, alors que le mésothéliome et le cancer de la vessie figurent dans les tableaux des maladies professionnelles, ils ne sont pas considérés comme directement liés à l’exercice du métier de sapeur pompier, car la liste des travaux susceptibles de les provoquer n’inclut pas l’extinction des incendies. Il revient donc aux intéressés eux mêmes de prouver ce lien, ce qui est souvent impossible en l’absence d’un suivi rigoureux de leur exposition. C’est dans ce contexte que cette proposition de loi prend tout son sens, puisqu’elle instaure un suivi systématique et uniformisé de l’exposition des sapeurs pompiers aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en rendant obligatoires l’élaboration et le renseignement d’une fiche d’exposition après chaque intervention à risque, intégrant notamment la composition des fumées. Ce dispositif, déjà encouragé par une circulaire émise par le ministère de l’intérieur en janvier dernier, doit aujourd’hui être gravé de la loi pour en garantir l’application effective et harmonisée sur l’ensemble du territoire. Il s’agit d’un outil essentiel pour améliorer la prévention, faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles et permettre une meilleure indemnisation des victimes. Protéger ceux qui nous protègent est un impératif, mes chers collègues. Cet enjeu dépasse les clivages politiques ; depuis des années, le Sénat s’est engagé sur cette question en légiférant et en travaillant au renforcement de la sécurité et de la reconnaissance des sapeurs pompiers. Je tiens à ce titre à saluer le travail des sénatrices Émilienne Poumirol et Anne Marie Nédélec, qui s’inscrit pleinement dans le prolongement de cet engagement. La mission d’information flash sur les cancers professionnels des sapeurs pompiers menée par nos collègues a mis en lumière une réalité trop longtemps ignorée ; elle a permis de souligner avec clarté et détermination l’urgence de renforcer la protection de ces femmes et de ces hommes qui, chaque jour, risquent leur santé pour assurer notre sécurité. Nous avons le devoir d’aller au bout de cette démarche et d’offrir aux sapeurs pompiers un cadre protecteur à la hauteur de leur engagement,

chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi transpartisane, portée par nos collègues Émilienne Poumirol et Anne Marie Nédélec, visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes,

Nos soldats du feu, professionnels comme volontaires, doivent apporter la preuve de la causalité professionnelle de la pathologie, une tâche ardue en raison de l’absence de fiches d’exposition aux facteurs de risque.

Cette évolution est conforme aux demandes exprimées par la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France (FNSPF). La transposition de ces dispositions dans la loi permettra de résoudre des difficultés récurrentes liées

il est des sujets intimes qui touchent au cœur même de notre pacte républicain et qui doivent à cet égard trouver un écho particulier au sein de nos assemblées parlementaires. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est avant tout l’expression d’une reconnaissance qui s’adresse à ceux qui, chaque jour, veillent à la sécurité des personnes, des biens et de notre environnement : aux sapeurs pompiers, mais aussi aux policiers, aux gendarmes et à tous ceux qui, dans l’ombre, protègent les plus vulnérables et garantissent nos libertés. Tous portent un uniforme qui symbolise bien plus qu’une fonction : un engagement, une mission, une exigence de chaque instant. La famille des sapeurs pompiers m’est particulièrement chère, car j’ai exercé en son sein pendant de pendant de très nombreuses années. Elle force l’admiration de tous et perpétue, jour après jour, les valeurs d’abnégation et de courage véritables, celles qui ne cherchent ni les honneurs ni les acclamations. pompiers braver les dangers, s’engager dans les flammes, affronter les catastrophes. Nous admirons tous la bravoure de ces femmes et de ces hommes, et nous connaissons leur dévouement sans faille. faille. Ce que nous voyons moins, ce que dissimule la grandeur de leur engagement, c’est l’usure que leur profession impose à leur corps : les souffrances invisibles qui s’accumulent et surgissent après des décennies, les substances toxiques et les fumées qu’ils inhalent, les particules fines qui s’insinuent dans leur peau, tous ces poisons chimiques qui s’infiltrent insidieusement dans leur

Comment accepter, mes chers collègues, qu’après avoir affronté le feu, le péril ou l’urgence, ils doivent encore lutter seuls pour faire reconnaître leurs blessures ? Est il acceptable de continuer d’infliger à leur dévouement sans faille l’épreuve supplémentaire du doute ? À ce stade, la gratitude, aussi sincère soit elle, ne suffit plus si elle ne s’exprime pas par des mesures de protection effectives. de protection effectives. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui constitue une indispensable avancée qu’il convient de saluer. Elle a pour objet l’établissement d’une fiche d’exposition obligatoire d’application nationale qui sera systématiquement renseignée par l’autorité territoriale, après chaque intervention à risque. Ce dispositif offrira enfin une traçabilité rigoureuse des substances auxquelles nos sapeurs pompiers sont exposés, garantissant ainsi une reconnaissance plus juste de leurs maladies professionnelles. là d’un changement attendu et nécessaire. Pourtant, mes chers collègues, aussi essentielle soit elle, cette loi, d’une certaine manière palliative, ne fait que répondre aux conséquences d’une situation déjà entachée. Il faut aller plus loin. Notre devoir ne se limite pas à reconnaître les maladies lorsqu’elles surviennent ; il est aussi, et surtout, de les empêcher d’apparaître. Ainsi, seule une politique de prévention ambitieuse sera à la hauteur de nos responsabilités et de leur engagement. Notre premier devoir est d’assurer une protection renforcée à nos sapeurs pompiers dès qu’ils affrontent le danger. Leurs équipements doivent être perfectionnés et leurs capacités à filtrer les substances toxiques renforcées

qui limitent l’exposition aux toxines, à l’image de certaines expérimentations menées en Seine Maritime.

Je tiens à saluer l’initiative de nos collègues Émilienne Poumirol et Anne Marie Nédélec, qui nous permettent aujourd’hui d’avoir ce débat très important, et à remercier madame la rapporteure de la commission des lois de son travail précieux sur ce texte. Mes chers collègues, nos sapeurs pompiers ne sont pas seulement les garants de notre sécurité ; ils sont les gardiens de nos valeurs. Ils interviennent sans distinction et sans condition. Ce texte ne concède ni faveur ni indulgence ; il rappelle simplement et sans ambiguïté à ces héros du quotidien que la Nation sait aussi protéger ceux qui la protègent. Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera à l’unanimité cette proposition de loi, mes chers

Cette proposition de loi de nos collègues Poumirol et Nédélec vise à améliorer la reconnaissance des cancers professionnels des sapeurs pompiers, ces derniers étant particulièrement exposés aux substances toxiques dégagées par les feux – des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques.

Cette proposition de loi apporte donc une première réponse pour améliorer la reconnaissance des cancers professionnels. Elle doit être complétée par le renforcement des actions de prévention, le rehaussement des protections des sapeurs pompiers et l’amélioration des réparations accordées aux

La mission sénatoriale souligne que « le développement d’équipements de protection individuelle adaptés aux risques se fait toujours attendre ». Elle préconise d’ailleurs le versement d’une dotation exceptionnelle aux Sdis pour acquérir des équipements de protection individuelle,

au delà de la reconnaissance des risques auxquels sont confrontés les sapeurs pompiers, au delà de l’ouverture des droits et des prises en charge auxquels ils doivent évidemment accéder, nous devons aussi les protéger, comme ils nous protègent au quotidien. La parole

qui nous proposent d’inscrire dans la loi les préconisations de leur rapport sur les cancers imputables à l’activité de sapeur pompier, ainsi que Françoise Dumont, rapporteure particulièrement investie sur ce sujet.

nous sommes à vos côtés. Pour autant, comme nous le rappelle cette proposition de loi, ces remerciements ne suffisent pas. Exposés à des produits de combustion dangereux, les sapeurs pompiers font face, du fait de leur activité, à des substances et à un niveau de risque qui a conduit le Centre international de recherche sur le cancer à classer, sans ambiguïté, cette activité comme « cancérogène pour l’homme ». Je prendrai un exemple : les PFAS, que les écologistes combattent de longue date. Les sapeurs pompiers étant largement exposés à ces substances dangereuses utilisées pour leurs propriétés

Face au risque probable d’une sous déclaration d’ampleur des maladies professionnelles des sapeurs pompiers, la construction des tableaux des maladies professionnelles doit être révisée au regard des dernières connaissances scientifiques. En France, seuls deux cancers sont reconnus comme des maladies professionnelles présumées chez les sapeurs

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction examen est le fruit d’un travail transpartisan, qui traduit notre capacité à transcender les clivages pour témoigner de notre attachement commun aux sapeurs pompiers, ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie au quotidien pour sauver celle des autres. Je tiens à saluer

Les risques liés à la profession de sapeur pompier doivent être pris en compte de manière concrète et efficace, au travers d’un suivi médical post professionnel et d’une reconnaissance des cancers imputables L’une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés est l’absence de données scientifiques fiables sur ces risques. En 2003, le rapport Pourny recommandait déjà la création d’une véritable veille sanitaire pour les sapeurs pompiers, notamment par la mise en place d’une banque nationale de données permettant de réaliser des études épidémiologiques. Hélas, aujourd’hui encore, aucun réel suivi médical coordonné n’existe et les études disponibles sont souvent contradictoires, ce qui empêche une prise en charge efficace.

qui met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi des risques professionnels, ainsi que des documents informatifs. Cette caisse finance en outre des études épidémiologiques qui alimentent la recherche médicale et scientifique. Depuis 2017, les fonctionnaires bénéficient d’une présomption d’imputabilité pour toute maladie inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, ce qui leur donne droit à des congés pour invalidité et au remboursement des frais médicaux.

En 2022, seules trente et une maladies professionnelles ont été répertoriées dans ce corps de métier. Ces chiffres faibles laissent penser qu’il existe une sous déclaration importante, probablement due aux difficultés pour prouver l’exposition, à l’absence de prise en compte de la polyexposition, ou encore à la complexité de la procédure de demande d’ATI. Cette situation entrave la traçabilité systématique des expositions et un suivi national uniforme de celles ci. Il est donc impératif de renforcer la prévention des risques,

En imposant la mise en place d’une fiche d’exposition pour chaque intervention, elle favorisera l’amélioration de la protection de nos sapeurs pompiers et facilitera la reconnaissance des maladies professionnelles.

diffusé sur l’excellente chaîne Public Sénat. Loin du cliché des héros infaillibles, ce film immersif évoque l’enjeu de la reconnaissance des maladies professionnelles de nos sapeurs pompiers, plus particulièrement des cancers causés par leur exposition répétée à des produits de combustion reconnus comme cancérogènes.

voire par ingestion, malgré les équipements de protection individuelle. En décembre dernier, dans cet hémicycle, le Gouvernement m’avait indiqué que le ministère du travail avait entamé

Par leur engagement sans faille à protéger, secourir et sauver, ils incarnent les plus belles valeurs de solidarité et d’humanité. Le Sénat, j’en suis sûre, poursuivra ses travaux pour continuer à les défendre et à les accompagner à leur juste valeur.

demande la parole ?… Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Belle

L’ordre du jour La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France, présentée par M. Pierre Jean Verzelen et plusieurs de ses collègues

Le problème, c’est qu’il s’en crée trop peu, notamment dans les communes rurales, à cause des contraintes administratives – les procédures, l’enquête publique, le recours à des cabinets d’études, etc. Tout cela prend du temps, coûte de l’argent, et c’est un frein. Nous proposons donc de ne plus recourir à l’enquête publique. En clair, si un maire souhaite restreindre le périmètre autour d’un édifice classé, il mène un travail en lien avec l’ABF ; puis une délibération du conseil municipal entérine cette Nous proposons de rendre publics et consultables en ligne les avis rendus par les ABF. Cela s’inscrit dans un mouvement global

est inspirée d’exemples réels de territoires qui se sont déjà organisés, de manière plus ou moins officieuse. L’idée est de créer, et de rendre obligatoire, un moment de dialogue et d’échanges sur les décisions qui sont rendues.

L’article 4, qui s’inscrit dans la droite ligne des travaux de la mission d’information, vise à tracer un cap, une orientation, et à mettre en avant le sujet de la réhabilitation en l’insérant dans la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, cher Laurent Lafon, monsieur

Pendant trop longtemps, la relation entre les architectes des Bâtiments de France et les acteurs locaux a souffert de trop d’incompréhensions. d’incompréhensions. Les ABF ont fait l’objet de critiques, de reproches, parfois au détriment de l’efficacité qu’exigent nos politiques patrimoniales, auxquelles nous sommes tous très attachés. Les ABF jouent un rôle fondamental.

Son ambition est simple : renouveler le dialogue entre nos architectes des Bâtiments de France et les acteurs locaux. L’article 1 vise ainsi à simplifier et à alléger les contraintes qui pèsent sur les porteurs de projet.

À l’article 2, il est proposé d’assurer la transparence des décisions rendues par les ABF, en prévoyant leur publication systématique dans un registre national. Depuis plusieurs années, nous sommes engagés dans un mouvement de transparence qui concerne tous les pans de l’action publique.

Ainsi, la rénovation respectueuse du bâti ancien, qui fait l’âme de nos communes, sera désormais un objectif partagé par tous les professionnels de l’architecture. Moins de contraintes, un meilleur dialogue et une ambition commune pour la réhabilitation : voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, le sens de cette proposition de loi. La ministre de la culture que je suis ne peut que se satisfaire de constater

et à la sauvegarde de nos cadres de vie. Les ABF y contribuent au quotidien. Avec cette proposition de loi, ils savent désormais qu’ils ne sont pas seuls. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France de notre collègue Pierre Jean Verzelen.

des acteurs clés tant pour ce qui concerne la préservation des sites protégés, l’aménagement du territoire, la valorisation de l’architecture et du patrimoine de nos territoires que pour la restauration des monuments historiques. Il en est toutefois de même de nos élus locaux, qui gèrent quotidiennement et directement les attentes des habitants et de l’ensemble des parties prenantes à l’aménagement du territoire dont ils ont la charge. La proposition de loi comporte quatre articles dont les objectifs sont les suivants : encourager la généralisation des périmètres délimités des abords ; assurer assurer la publicité des décisions rendues par les ABF ; renforcer le dialogue entre les élus, les porteurs de projet et les ABF ; et enfin, ériger la réhabilitation du bâti ancien en priorité partagée par tous les acteurs concernés. Le recours aux périmètres délimités des abords permettra notamment aux élus locaux d’adapter les limites des zones de protection des monuments historiques aux réalités locales.

le terrain. L’article 1 du présent texte vise à remédier à cette situation, en favorisant la généralisation des PDA. L’article 2 rend obligatoire la publicité des avis rendus par les ABF et prévoit la publication systématique de leurs décisions dans un registre national accessible en ligne pour le public. Nous saluons cette mesure

Enfin, l’article 4 modifie la loi du 3 janvier 1977 en ajoutant la réhabilitation des constructions existantes au champ de l’intérêt public associé à l’architecture. L’enjeu est simple : inscrire dans le droit le fait que la réhabilitation relève d’un objectif partagé par tous les professionnels de l’architecture, afin d’éviter les pratiques délétères pour le bâti ancien.

cet équilibre. Je tiens à saluer ce travail, nourri des propositions issues de la mission d’information relative au périmètre d’intervention et aux compétences des architectes des Bâtiments de France, à laquelle j’ai eu la chance de participer. Cette mission d’information est partie du constat d’une forme d’incompréhension entre les ABF et certains élus locaux ou porteurs de projets.

Cette mission d’information a réuni des sénateurs issus de différentes commissions et de différentes obédiences politiques, aux points de vue très éloignés les uns des autres. Certains espéraient même pouvoir, grâce à cette mission, remettre en question les principes fondamentaux de la protection patrimoniale.

se réunira périodiquement pour examiner les dossiers ayant reçu un avis défavorable ou un avis favorable assorti de trop lourdes prescriptions. La proposition de loi ajoute enfin la réhabilitation des constructions au champ de l’intérêt public associé à l’architecture. Il sera certainement utile de débattre ultérieurement de la nécessité d’associer les architectes plus en amont des projets de réhabilitation, afin de lutter contre les interventions inadaptées sur le bâti patrimonial non protégé.

Elle fait l’objet d’un large consensus, ce qui lui vaut d’être inscrite dans un espace transpartisan. Ce texte constitue la traduction législative des recommandations formulées dans le rapport de la mission d’information

ces travées, nombre d’entre nous ont été associés aux travaux des ABF et des élus dans nos départements respectifs. Nous avons ainsi été les témoins des incompréhensions mutuelles et des frustrations que les avis rendus peuvent parfois susciter.

de la proposition de loi est ainsi de « renouveler les conditions du dialogue entre les ABF, les élus locaux et l’ensemble de nos concitoyens ». Le texte prévoit en premier lieu de simplifier le recours aux périmètres délimités des abords des monuments historiques, afin de favoriser leur généralisation.

pertinents sur le papier et qu’ils sont sollicités tant par les élus que par les ABF, leur création se heurte à des lourdeurs administratives souvent décourageantes. Seuls quelques milliers d’entre eux ont vu le jour depuis leur création, alors que l’on compte près de 45 000 monuments historiques dans notre pays. Pour faciliter le travail des communes, notamment

obligatoires. Nous partageons l’objectif de permettre aux conseils municipaux de se saisir davantage des politiques de conservation du patrimoine, avec l’aval des ABF.

En renforçant le dialogue pour concilier les enjeux patrimoniaux et environnementaux, ce texte vise à rendre l’action des ABF plus lisible et à mieux l’adapter aux réalités locales. La mission d’information, à laquelle notre collègue Guylène Pantel a participé, a mis en évidence plusieurs points de friction qu’il nous appartient aujourd’hui de corriger.

Enfin, concilier protection du patrimoine et rénovation énergétique du bâti reste un défi majeur, surtout pour l’isolation des bâtiments anciens et l’installation de panneaux photovoltaïques. divers blocages appellent des réponses concrètes pour garantir la compréhension des décisions et leur meilleure adaptation aux réalités locales. Il ne s’agit ni de déposséder les architectes des Bâtiments de France de leur rôle ni de sacrifier notre patrimoine sur l’autel de la modernité. Il s’agit d’introduire davantage de souplesse et de concertation, afin d’adapter le cadre réglementaire aux besoins concrets des territoires. En Gironde, par exemple, de nombreux projets de rénovation et de réhabilitation se heurtent à des refus ou à des demandes de modifications

Elle simplifie la procédure de création des périmètres délimités autour des monuments historiques et permet aux élus d’instaurer un règlement encadrant l’architecture et l’esthétique des constructions dans ces zones sensibles. par ailleurs la publication systématique des avis des ABF sur une plateforme en ligne. Aujourd’hui, ces décisions restent trop peu accessibles, ce qui alimente un sentiment d’opacité. autre avancée significative. Trop souvent, les projets se heurtent à des refus mal compris, entraînant des recours longs et coûteux. Cette instance offrira un cadre de dialogue adapté pour aboutir à des solutions partagées. Nous considérons néanmoins que les élus locaux doivent être pleinement associés à ces échanges. Tel est le sens de l’amendement n° 1 rectifié, que notre collègue Guylène Pantel défendra à l’article 3. Mes chers collègues, l’examen de cette proposition de loi nous rappelle que la protection du patrimoine et l’innovation sont les deux faces d’une même pièce. Ce texte modernise un cadre parfois trop rigide, tout en garantissant la transmission des trésors architecturaux qui font la richesse de nos territoires, sans remettre en cause l’avis conforme, acquis inestimable de notre droit, auquel l’ensemble de la commission de la culture est attaché.

L’article 2, quant à lui, a pour objet d’améliorer la transparence des avis rendus par des ABF, en prévoyant leur publication systématique dans un registre national numérique mis à disposition du public. L’article 3 instaure une commission départementale chargée de l’examen collégial des dossiers litigieux et de ceux qui pourraient le devenir. Dans sa recommandation n° 1, la mission d’information préconisait de créer une commission départementale pour favoriser la conciliation le plus en amont possible,

patrimoine), que nous connaissons bien. Oui ! Plus d’ABF, c’est plus de temps sur le terrain, plus de temps pour négocier, concilier, expliquer, bref, plus de temps pour faire apprécier –

Cette discussion aura donc lieu de nouveau dans cette enceinte, à l’autonome prochain. Je vous donne rendez vous, madame la ministre ! Très bien Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la qualité de l’architecture de notre quotidien et la préservation du patrimoine bâti sont des politiques menées de longue date par le ministère de la culture. Elles constituent le fondement de son action publique et sont célébrées comme constitutives de l’identité culturelle de notre pays. Cependant, elles sont également trop souvent la source de tensions entre les élus et l’État, l’intervention de ce dernier étant parfois considérée comme une entrave à la liberté de construire.

maires, et des tracasseries bureaucratiques liées aux autorisations d’urbanisme. Il est donc crucial de rendre hommage à leur travail, à leur dévouement et à leurs efforts sincères pour tenter de concilier les obligations imposées par une législation protectrice et les souhaits souvent contradictoires des pétitionnaires et des autorités chargées de délivrer les permis. le, les maires n’ont aucun intérêt à un affaiblissement de l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France, car cela les exposerait à des contentieux actuellement assumés par l’État.

contre les avis des ABF. Partout où un dialogue constructif s’est instauré entre les services des ABF et ceux de la collectivité qui sont chargés de l’urbanisme, les conflits sont rares et résolus par la négociation. En revanche, des différends peuvent surgir lorsque les ABF peinent à assumer pleinement leur mission de conseil auprès d’élus de communes démunis face à la complexité du droit du patrimoine. Ce constat n’est pas nouveau. Dans un rapport remis en octobre 2018 à la ministre de la culture, M. Philippe Bélaval, aujourd’hui conseiller du Président de la République, faisait cette mise en garde

à donner une priorité, dans la répartition de leur temps, aux avis, débouchant sur une restriction de l’exercice de leurs autres compétences. Le déséquilibre ainsi créé est fâcheux en enfermant trop les Udap dans un rôle d’empêchement, il pèse très négativement sur l’image, non seulement des architectes des Bâtiments de France, mais aussi des dispositifs de protection eux mêmes en outre, il affaiblit le rôle que le ministère de la culture est susceptible de jouer sur les territoires pour la préservation d’un cadre de vie de qualité. » Sur le fondement de cette analyse, toujours d’actualité, vous aviez, madame la ministre, proposé dans votre plan présenté en juillet 2024, intitulé Printemps de la ruralité,

L’architecture impose une immersion totale. Ce n’est pas comme composer de la musique ou écrire une comédie. […] Une musique laide, on peut ne pas l’écouter ; un tableau laid, on peut ne pas le regarder, mais un immeuble laid reste là, devant nous, et nous sommes bien obligés de le voir. Ces quelques mots d’avertissement de l’architecte Renzo Piano justifient à eux seuls les missions des architectes des Bâtiments de France : veiller à ce que les lubies immobilières de quelques uns ne défigurent pas les perspectives architecturales du plus grand nombre.

Les dispositions de la proposition de loi permettront de répondre aux deux premières critiques. Les travaux de la mission d’information sur les ABF auront permis de démystifier les conditions d’exercice de leurs compétences. Nos auditions ont en effet permis de comprendre que, au regard de l’ensemble des avis, le taux de refus est assez faible, En outre, une décision défavorable ne fait pas totalement obstacle à un projet, car elle peut toujours donner lieu à un échange. Ainsi, en définitive, seulement 0,1 % des projets seraient refusés, ce qui conduirait à moins d’une dizaine de contentieux par an. est très faible en comparaison du contentieux de l’urbanisme et de l’aménagement porté devant les tribunaux administratifs – 12 700 affaires jugées en 2024 – ou du contentieux de la construction porté devant le juge judiciaire – 33 500 affaires en 2024.

Elles instaurent un peu de flexibilité, avec la généralisation des périmètres délimités des abords, et une meilleure compréhension de la « jurisprudence » des ABF, grâce à la publicité des avis.

Pourtant, il existe des exemples à l’étranger. L’Italie offre une piste intéressante pour concilier conservation, rénovation et production d’énergie renouvelable

Je tiens à remercier nos collègues d’avoir pris en considération la nécessité d’inscrire la notion de réhabilitation dans la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Choisir de réhabiliter plutôt que de démolir permet de préserver les ressources naturelles, de réduire les déchets et les émissions de CO2 et d’optimiser l’empreinte écologique de nos milieux habités. Réhabiliter, ce n’est pas seulement rénover, restaurer et mettre aux normes ; c’est un travail subtil de transformation, par lequel l’acte architectural permet de conjuguer mémoire, performance et usage. Aujourd’hui, la beauté de nos territoires urbains et ruraux peut être mise en danger par des constructions court termistes. Dans la Grèce antique, les élus athéniens commençaient leur mandat par ce serment Je vous promets, Athéniens, de vous rendre Athènes plus belle que vous me l’avez donnée. » L’architecture participe au bien être de nos concitoyens, renforce le désir d’appartenir à une société.

Les architectes des Bâtiments de France, qui œuvrent au quotidien pour assurer la préservation de notre patrimoine et de notre cadre de vie, sont les précieux gardiens de ce récit commun. Il suffit, pour en avoir la certitude, de se promener dans les si belles rues d’une commune comme Figeac, exemple souvent cité de coopération efficace entre ABF et élus. Son architecture attire chaque année, dans le département du Lot, des centaines de milliers de touristes venus du monde entier. Nous le savons, néanmoins, le rôle des architectes des Bâtiments de France a parfois suscité des débats au sein de notre hémicycle.

est une illustration parfaite, à mon sens, des consensus auxquels peut parvenir le Sénat. Partis de positions initiales parfois divergentes, nous avons su aboutir, à l’issue d’un travail rythmé – vingt auditions, quatre déplacements, 1 500 témoignages d’élus locaux –, à des propositions communes, nourries par une approche pragmatique collant au plus près du terrain. Il en est ressorti plusieurs mesures d’ordre législatif, encore affinées par le travail du rapporteur, qui a tenu à faire un nouveau tour d’horizon des acteurs clés concernés par leur mise en application. L’article 1 du texte encourage la généralisation des périmètres délimités des abords. Ces périmètres, dits intelligents, créés par la loi de 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, avaient pour vocation de rationaliser la protection patrimoniale aux abords des monuments, afin de limiter l’intervention des ABF aux emplacements où la covisibilité fait consensus.

et de la conserver dans les cas où le PDA étend le périmètre de la protection au delà de 500 mètres. Afin d’améliorer la prévisibilité des décisions prises par les ABF, cet article permettra également aux élus qui le souhaitent d’élaborer un règlement du PDA en lien avec l’ABF. La rédaction initiale prévoyait que ce règlement serait autonome, autonome, dans un souci de rationalisation des outils réglementaires ; finalement, il est prévu que le règlement du PDA s’inscrira dans le plan local d’urbanisme. L’article 2

par le plus grand nombre. L’article 3 crée une commission de conciliation permettant un examen collégial des dossiers, afin de favoriser l’émergence de solutions concertées sur les dossiers les dossiers litigieux, avant l’engagement de procédures de recours. Il s’agit de généraliser à l’ensemble du territoire national de bonnes pratiques qui existent déjà dans certains départements, où se réunissent, sur l’initiative du préfet, ABF, maires et porteurs de projet, afin de lever, par le dialogue, les difficultés rencontrées en amont de la procédure de recours. Cette mesure a suscité de nombreuses interrogations de la part des acteurs entendus en audition, ce qui a conduit à une réécriture significative du dispositif par le rapporteur, notamment pour préciser sa composition et son articulation articulation avec la procédure de recours. Enfin, l’article 4 ajoute à la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture la notion de réhabilitation, afin d’intégrer celle ci parmi les activités architecturales d’intérêt public, dans le dessein de répondre à la préoccupation de faire de la réhabilitation du bâti ancien un objectif partagé par l’ensemble des acteurs du secteur de la rénovation. C’est une dynamique déjà amorcée, qu’il convient d’encourager. Je tiens pour conclure à souligner que, tant lors des travaux de la mission d’information que pendant les auditions préparatoires à cette proposition de loi, la problématique du manque de moyens humains et d’ingénierie dans les territoires pour pour préserver notre patrimoine a été abondamment soulignée. Je l’ai moi même rappelée lors de l’examen du budget, au moment où le Sénat a adopté un amendement visant à recruter un ABF supplémentaire par département. Nous ne pouvons éluder ce sujet si nous voulons diminuer de façon significative leur charge de travail d’augmenter le temps qu’ils consacrent à leurs missions de conseil et d’accompagnement. Les sénateurs et sénatrices socialistes voteront en faveur de ce texte, qui s’inscrit pleinement dans la continuité de la mission d’information dont il est issu

les ABF sont confrontés à l’inflation patrimoniale des dernières décennies et à l’élargissement progressif des espaces protégés. À l’image du dieu Janus, ayant une face tournée vers le passé et l’autre vers l’avenir, les ABF – les « acteurs de la beauté de la France

côté, le dialogue confiant, exigeant et permanent de notre ancien collègue sénateur Yves Dauge, alors président de sa communauté de communes rurales, avec le service départemental d’architecture a permis, au prix d’une patiente pédagogie, d’entraîner les neuf maires concernés à préserver et à protéger le patrimoine et les paysages ruraux du pays de Rabelais,

de loi contient des évolutions positives, telles que la généralisation des périmètres délimités des abords, qui permettra une approche plus fine des protections à opérer, ou la publication des décisions rendues par les ABF, afin d’objectiver en toute transparence les motivations de leurs décisions.

Si sa composition, qui devra rester limitée, est à l’image de celle de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ses membres seront éclairés, assidus, et permettront, à mon avis, de résoudre Toutefois, ces avancées législatives ne régleront pas tous les problèmes des relations des ABF avec les maires et nos concitoyens. Il conviendrait aussi, à mon avis, comme cela a été évoqué lors de la visite de notre commission à la Cité de l’architecture et du patrimoine au palais de Chaillot, que la formation des ABF intègre un module sur la vie et la gestion locales, afin que les étudiants s’imprègnent des contraintes des maires, notamment en milieu rural.

Ces guides et ces référentiels doivent être travaillés en liaison étroite avec les collectivités. Ils doivent avoir des déclinaisons départementales adaptées aux territoires et travaillées conjointement avec les services de l’État,

dans leurs interactions avec les institutions. C’est pourquoi je propose de remplacer l’enquête publique par une consultation du public par voie électronique. Cette démarche permettrait de réduire les coûts administratifs, de renforcer la participation citoyenne et de simplifier le traitement des observations recueillies. Avec votre soutien, mes chers collègues, nous œuvrons en faveur d’une administration plus moderne, plus proche des citoyens et plus respectueuse de leurs attentes.

Mme Catherine Belrhiti. Cet amendement, qui me semble essentiel, vise à harmoniser les pratiques des architectes des Bâtiments de France dans le cadre de leur mission de contrôle, par la création d’un document référentiel national, élaboré par une commission d’experts et centralisant un ensemble un ensemble de critères d’intervention standardisés. Cette initiative est une réponse à une inquiétude croissante : nombreux sont les élus et les porteurs de projet qui déplorent l’imprévisibilité et l’incohérence des décisions rendues par les ABF, lesquelles varient d’un département à l’autre. La protection de notre patrimoine commun doit répondre à des objectifs partagés. Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir cet amendement qui permettra de guider les ABF dans leur mission de contrôle et d’assurer une application homogène des normes sur notre territoire. Pas bête ! Quel

sera celui de la commission de conciliation, si l’on daigne y accorder aux maires une place centrale et décisionnelle. À l’heure actuelle, les architectes des Bâtiments de France sont trop souvent un frein

pour examiner le dossier après réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. L’objectif est de garantir une réelle concertation entre les différentes parties prenantes, notamment les élus locaux, les services de l’État et les experts du patrimoine. Un délai d’un mois apparaît trop contraint au regard des enjeux soulevés par les projets concernés et de la nécessité d’une instruction approfondie. La mise en œuvre d’un recours dans un délai d’un mois pose une difficulté au regard des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. Pour un permis de construire, l’architecte des Bâtiments de France dispose de deux mois pour rendre son avis, et la durée totale d’instruction est de trois mois maximum. Créer une commission départementale

Nos élus locaux, entrepreneurs, associations et particuliers nous le disent, dans les territoires, régulièrement : ils désirent un dialogue direct, constructif et réactif avec le corps des architectes des Bâtiments de France.

de département ou son représentant, l’ABF ou son représentant, les représentants des associations d’élus, le pétitionnaire et le maire de la commune concernée par le dossier – voilà le bloc de base. Il est indiqué que cette liste est non exhaustive et que le préfet peut y inviter les associations patrimoniales, le CAUE,

Belrhiti. Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commission de conciliation dans le processus décisionnel en lui conférant le pouvoir d’émettre un avis conforme

que les élus locaux ont souvent le sentiment d’être confrontés à des avis et à des injonctions contradictoires : on leur dit qu’il ne faut plus artificialiser – cet objectif, nous le partageons

à isoler leur bien par l’extérieur avec des matériaux inadaptés, provoquant des dégâts irréversibles sur des constructions traditionnelles, notamment celles qui comportent du bois en façade. Ces travaux, de surcroît, dénaturent l’identité visuelle du

de modifier l’article 1 de la loi de 1977 sur l’architecture, qui ne vise actuellement que les permis de construire, pour y inclure toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, c’est à dire les permis de construire, les déclarations préalables, les permis de démolir, les permis d’aménager.

font du patrimoine de la France ce qu’il est.